énumérés par le code de l'urbanisme, qui renvoie aux dispositions générales sur les objectifs des politiques d'aménagement. Parmi ces motifs, on compte la mise en oeuvre d'un projet urbain ou d'une politique locale de l'habitat, l'organisation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la réalisation d'équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, le renouvellement urbain, enfin, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. naturels. Rien dans cette liste ne permet aux élus d'agir à titre préventif pour la maîtrise de leur territoire en luttant contre la flambée des prix et, notamment, la spéculation immobilière. Plusieurs délibérations municipales ont d'ailleurs été censurées parce qu'elles évoquaient la lutte contre la spéculation foncière pour justifier du droit de préemption, alors que d'autres délibérations ont pu être acceptées, parce qu'elles contournaient les différents méandres du contrôle de légalité.

Sa vocation est d'accompagner ses adhérents dans le portage foncier, afin de développer la construction du logement social et l'activité économique. Depuis sa création, en 1996, le syndicat a porté un total de 285 millions d'euros de foncier, permettant l'aboutissement de dizaines de projets d'aménagement urbain sur l'ensemble du Val-de-Marne. Ces projets sont le fruit d'un partenariat constant et de proximité entre le syndicat, les communes, le département, les offices publics d'habitat social, les sociétés d'économie mixte, les établissements publics d'aménagement et l'EPF d'Île-de-France. Le SAF 94 intervient aujourd'hui aux côtés de plusieurs communes carencées- Le Plessis-Trévise, Marolles-en-Brie, Noiseau, Périgny-sur-Yerres -, les accompagnant dans la constitution de réserves foncières en vue de réaliser des opérations de logements sociaux. La délégation du droit de préemption urbain par les services de l'État est donc nécessaire pour que se poursuivent ces interventions foncières. C'est ainsi que l'on garantira la bonne réalisation de ces projets de construction et que l'on poursuivra le développement de nouveaux programmes de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU.

puisse le déléguer à tout établissement public y ayant vocation. Toutefois, l'article visé par cet amendement, qui concerne les communes « carencées », ne le précise pas expressément. Sur ce point juridique, la commission demande l'avis du Gouvernement.

à la réserve foncière. Certes, les établissements publics fonciers existent, mais on voit bien que leur capacité à intervenir dépend de la capacité à libérer du foncier.

qui ont eu cours dans mon département, dans des communes que nos collègues du groupe CRCE connaissent assez bien. Comme cela a été exposé sur la place publique, je vais brièvement rappeler ce qui se passait. Les maires convoquaient les promoteurs, pour lutter contre la spéculation, et leur disaient : « Écoutez, monsieur, si vous voulez un permis de construire, on vous interdit de vendre à plus de tant du mètre carré.-

principe de ce dispositif est de permettre aux communes d'être informées quand il y a vente à la découpe ou congé pour vente et que les locataires ne peuvent pas accepter la vente du logement qui est ainsi mis sur le marché.

donc que la formulation du présent amendement répond aux injonctions du Conseil constitutionnel, tout en reprenant une idée qui est importante, puisque l'on sait que, dans certains cas, ces congés pour vente déstabilisent considérablement des locataires fragiles.

Force est de constater que votre amendement tend à restaurer des dispositions très similaires à celles qui ont été déclarées inconstitutionnelles. Votre rédaction modifie simplement la formulation relative à l'objectif de garantie du maintien dans les lieux des locataires

Par cet amendement, nous nous attachons particulièrement aux conséquences de la hausse exponentielle des prix du foncier Concrètement, aujourd'hui, les collectivités ou organismes qui veulent intervenir en matière de construction de logements publics doivent au préalable acquérir des terrains, acquisition qui pèse entre 14 % et 25 % du coût global du programme de construction. Pour ce faire, les collectivités disposent de deux outils : le droit d'expropriation, dispositif largement encadré, et le droit de préemption. Pour autant, la mise en oeuvre de ces instruments est soumise à l'évaluation du service des domaines, qui détermine le prix d'acquisition en se fondant sur les prix de marché. Or, comme nous l'avons déjà souligné, ceux-ci connaissent une hausse exponentielle en zone dense ou touristique. ou touristique. Pour éviter les surcoûts fonciers dans le cadre d'opérations d'aménagement d'utilité publique, il convient donc de mettre en oeuvre un mécanisme permettant de fixer le coût du foncier au jour de la définition d'un périmètre d'opération révisé suivant l'inflation à l'indice de la construction. Il s'agit de poser en quelque sorte un principe d'absence d'enrichissement sans cause. En effet, aujourd'hui, lorsque la collectivité définit un périmètre de projet d'aménagement, la valeur du foncier situé sur ce périmètre augmente fortement, du fait même de l'existence de ce projet. Quand on sait le temps que peut mettre une opération à sortir de terre, nous devinons aisément que les surcoûts fonciers peuvent être exorbitants ! Cette situation pernicieuse conduit à faire payer par les collectivités la plus-value foncière résultant de leur volonté d'aménagement. Il ne s'agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs. Il convient seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l'immobilier, permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités à définir une programmation d'acquisition des terrains à bâtir, nécessaire à la construction de logements accessibles à tous.

Les voies situées dans des zones d'activités ou commerciales sont, pour le moment, exclues du dispositif permettant de transférer la propriété des voies privées dans le domaine public sans indemnité, à la suite d'une enquête publique.

Cet amendement a pour objet de libérer des capacités de construction et de ne pas pénaliser les collectivités oeuvrant pour la mixité fonctionnelle. Il serait donc opportun d'étendre l'application de l'article L. 318-3 du code de

toujours un fléau lancinant, récurrent et bloquant, à savoir que l'État ne perçoit pratiquement rien sur les actifs successoraux et sur les dévolutions successorales qui ne se font pas, car l'on n'arrive pas à faire la répartition, les co-indivisaires étant parfois difficiles à trouver. On a inventé un dispositif à Mayotte jusqu'en 2028, qui consiste à assainir le cadastre et à régler, si j'ose dire, le désordre des propriétés.

Certes, on peut dire que, par imitation et par répétition, on veut voir appliquer dans les outre-mer ce qui se pratique depuis quelque temps en Corse,

fiscal, cela ne marchera pas. Au-delà de l'unanimité émise sur un texte de bon aloi et équilibré, sans cet accompagnement fiscal sur les droits de mutation et sur les droits de succession, y compris ce que l'on appelle le cantonnement, on ne sortira pas du désordre des propriétés.

Le projet de loi veut encourager la transformation des bureaux vacants en logements. Nous sommes favorables au « bonus de constructibilité » de 30 %, c'est-à-dire à des droits à construire supplémentaires. En revanche, l'article 9 permettra également de passer outre les obligations de mixité sociale prévues par les plans locaux d'urbanisme, sauf dans les communes carencées en logements sociaux. Les servitudes de mixité sociale intégrées dans les PLU traduisent une volonté politique des élus de favoriser la production de logements sociaux sur leur territoire. Permettre cette dérogation n'a donc aucun sens. Par ailleurs, c'est considérer que la réalisation de logements sociaux est un frein à la production de logements. Ce type de raisonnement n'est plus acceptable dans un pays qui manque de logements à des prix abordables pour la plupart des Français. Les mesures incitatrices pour transformer les locaux de bureaux en logements ne doivent pas se faire au détriment du logement social et de la mixité. Il s'agit donc de supprimer cette dérogation.

que je ne peux que partager. Rappelons que le stock de bureaux non utilisés était évalué à près de 3,5 millions de mètres carrés en Île-de-France, en 2017. Toutefois, Toutefois, pour atteindre cet objectif, est accordée la possibilité de déroger aux servitudes de mixité sociale prévues par les PLU, sauf dans le cas des communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence. Cette disposition nous semble contraire aux objectifs de mixité sociale et à l'esprit de la loi SRU. En effet, les communes carencées ne représentent qu'une partie des communes qui sont en dessous des 25 % de logements sociaux. Elles invoquent souvent, comme justification de cette situation, le manque de foncier pour construire des logements sociaux. Or la transformation de bureaux permettrait bien de dégager des espaces pour construire des logements sociaux dans ces zones tendues. Cet amendement vise donc à réintroduire la servitude de mixité sociale dans le cadre des opérations de conversion de bureaux en logements. L'amendement

Ces locaux sont bien plus utiles en étant transformés en logements, plutôt qu'en restant à l'abandon. Pour autant, nous contestons le fait que, pour faciliter cette conversion, il soit permis de déroger aux règles de mixité sociale définies dans le cadre du plan local d'urbanisme. L'objectif de mixité sociale constitue une valeur primordiale de cohabitation sociale dans nos sociétés démocratiques, induisant un impératif de « vivre ensemble ». S'il semble raisonnable de déroger à des règles de hauteur ou de gabarit tenant à la structure même du local, renoncer aux ambitions en matière de mixité sociale ne semble pas acceptable. Cet amendement vise donc à réintroduire l'obligation du respect de l'exigence de mixité sociale pour les dérogations au PLU, permise par le présent article, pour les communes ayant un fort enjeu de densification, et de réponse aux besoins de logement. de cet amendement permettrait de faire de cet « objectif de mixité sociale » une condition non négociable, en la prévoyant pour l'ensemble des cas de figure indiqués à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, qui énonce les possibilités de dérogations au PLU. Quel

Je rappelle que la dérogation accordée dans le projet de loi ne remet absolument pas en cause la volonté des élus de promouvoir la mixité sociale dans leurs plans locaux d'urbanisme. De plus, la dérogation vise non les constructions nouvelles, mais la transformation de bureaux en logements. Les prescriptions du PLU continuent à s'imposer aux autres projets, y compris à l'échelle des programmes, et la décision d'accorder ou non cette dérogation est bien prise par le maire. Par conséquent, les servitudes de mixité sont toujours applicables à l'échelle de la commune. Cette dérogation encadrée reste un outil

est ainsi libellé : La parole est à M. Fabien Gay. Pour prolonger nos débats sur la question des bureaux vacants, nous voulons aborder la question des logements vacants, par le renforcement de la taxe qui affecte ses logements en zones tendues, marquées par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Nous reprenons en réalité une proposition formulée par la Ville de Paris, le 17 juin 2017, dans un voeu du conseil municipal. Il y a environ 100 000 logements vacants

Le 15 décembre 2016, une taxe sur les logements vacants, la TLV, a été créée. Je rappelle qu'elle ne concerne que les villes de plus de 50 000 habitants où existent des difficultés d'accès au logement. Le montant actuel de cette taxe à Paris, par exemple, est en moyenne de 1 000 euros la première année et de 2 000 euros la deuxième année, ce qui représente 12,5 % de la valeur locative du bien la première année et 25 % la deuxième

-contre la vacance spéculative. Il n'est pas concevable qu'il soit aujourd'hui plus rentable pour certains propriétaires de conserver des logements vacants plutôt que de les mettre sur le marché. Il est donc nécessaire, comme nous le proposons, d'augmenter la taxe sur ces logements vacants.

Il s'agissait de créer des places de logement temporaire dans des locaux vacants, mis à disposition par leurs propriétaires, qui s'assuraient ainsi de leur préservation. Le présent article, inséré à l'Assemblée nationale, revoit totalement cette possibilité en l'orientant exclusivement vers l'hébergement.

créant un bail dégradé et absolument pas protecteur. Nous proposons donc, puisque l'expérimentation n'a pas été concluante pour le logement, de maintenir l'orientation de ce dispositif exclusivement vers l'hébergement, seule manière de le rendre acceptable.

dit, il y a une grande différence entre l'hébergement et le logement, même si le logement est temporaire. C'est pourquoi j'émettrai un avis défavorable sur votre amendement. Quand vous occupez un logement, vous avez une adresse, et cela change tout.

c'est-à-dire en cours de changement d'usage. Le constat est simple : plus de 145 000 personnes dorment aujourd'hui dans la rue ; 1,8 million de demandeurs de logements sociaux attendent une proposition de logement social, parfois depuis plusieurs années.

Dans chaque département en secteur tendu serait mise en place, sous la responsabilité du préfet, une commission intégrant les opérateurs associatifs du logement et de l'hébergement du territoire. Elle serait intitulée « commission de mobilisation des bâtiments vacants pour répondre à l'urgence sociale de cette commission serait d'étudier la création de structures d'hébergement ou de logements pendant la durée de la vacance intercalaire. Ainsi, chaque mise en vacance d'un bâtiment appartenant à des collectivités territoriales, des établissements publics, à des bailleurs sociaux ou à l'assistance publique, un signalement devrait obligatoirement être réalisé auprès de cette commission.

Dans le même temps, plus de 145 000 personnes dorment dans la rue et 1,8 million de personnes attendent un logement social. Vous pouvez imaginer les conséquences sociales, humaines et économiques de cet état de fait. Il y a donc bien une urgence sociale. Qu'ils soient la propriété de l'État, des collectivités, des bailleurs sociaux, des établissements publics ou de l'Assistance publique, les bâtiments inoccupés sont nombreux et les raisons de cette vacance, multiples : changement d'affectation, bâtiments en attente d'un projet ... L'État doit être exemplaire sur cette question. Cet amendement vise donc à mieux identifier et à mieux mobiliser ce patrimoine, qualifié d'« intercalaire ». Dans chaque département en secteur tendu, et sous la responsabilité du préfet, une commission intégrant les opérateurs associatifs du logement et de l'hébergement du territoire pourrait être mise en place. Dénommée « commission de mobilisation des bâtiments vacants pour répondre à l'urgence sociale », elle serait chargée d'étudier la création de structures d'hébergement ou de logement pendant la durée de la vacance intercalaire. À chaque mise en vacance d'un bâtiment appartenant à des collectivités territoriales, à des établissements publics, à des bailleurs sociaux ou à l'assistance publique, un signalement devrait obligatoirement être réalisé auprès de cette commission.

avons pris des engagements très clairs : 40 000 intermédiations locatives, 10 000 pensions de famille, 40 000 logements dits « adaptés », auxquels s'ajoutent 20 000 logements vacants pour les personnes réfugiées.

Il est vrai que les gouvernements, quels qu'ils soient, sont face à ce problème d'urgence et la seule façon d'agir efficacement, c'est de travailler directement avec le préfet, ... Voilà ! ... et que celui-ci agisse directement en partenariat avec les collectivités locales. Le préfet ne peut rien faire

que ce n'est pas en créant une commission supplémentaire qu'on résoudra ce problème, et je vous le dis très clairement. Elle peut

Le scrutin est ouvert.

nécessaire. Je veux rassurer le législateur quant à l'application pragmatique des dispositions. D'une part, le code pénal précise que l'annulation d'une disposition réglementaire postérieurement à l'édification de l'ouvrage ne peut conduire l'autorité judiciaire à constater une infraction, faute de pouvoir démontrer, par la force des choses, un élément intentionnel. intentionnel. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue. Au moment de la construction de l'ouvrage, le constructeur qui respecte l'état du droit en vigueur ne peut pas avoir conscience, par définition, de commettre une infraction. D'autre part, le juge administratif peut apprécier les conséquences des effets rétroactifs de l'annulation d'un acte réglementaire. Il est même en capacité de déroger au principe de l'effet rétroactif. Dans ce cas, l'autorité judiciaire saisie d'un constat d'infraction est amenée forcément à classer sans suite. Par conséquent, il n'y a, selon moi, aucune difficulté. Je comprends que la question soit posée, car ce

pour l'attributaire de logements et de bureaux vacants réquisitionnés pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri, de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. Il s'agit également de maintenir la même durée de la réquisition, sans avoir à distinguer entre l'hébergement d'urgence et les autres cas de réquisition.

Le projet de loi prévoit que les locaux réquisitionnés pour accueillir de l'hébergement d'urgence peuvent faire l'objet de « travaux de mise aux normes minimales requises en fonction de l'usage prévu pour les locaux en lieu et place de la mention « travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité ». Or nous savons bien ce qu'il en est des normes applicables en fonction de l'usage. La France s'est engagée sur l'amélioration des conditions d'accueil en centres d'hébergement. Le rapprochement entre les normes minimales de décence en hébergement et celles qui dont en vigueur dans le logement est défendu depuis 2009, notamment dans le cadre du programme d'humanisation des centres d'hébergement. L'individualisation des chambres et des sanitaires, par exemple, est considérée par l'ensemble des acteurs comme fondamentale, comme un préalable à tout accueil respectueux de la dignité des personnes. Elle permet aux résidents de bénéficier d'un espace d'intimité et de liberté essentiel à leur bien-être et garantit une meilleure qualité d'hygiène. Cette ambition doit rester prioritaire pour sortir des logiques de simple mise à l'abri des personnes en situation de précarité. C'est d'ailleurs un objectif que les députés ont traduit dans d'autres dispositions du projet de loi, notamment à l'article 43 consacré à l'amélioration de la prise en charge des personnes sans domicile fixe. Enfin, faut-il le rappeler, la durée moyenne en centres d'hébergement se situe autour de quatorze mois, mais il peut arriver que certaines personnes restent plusieurs années dans les centres d'hébergement. Cet amendement a donc pour objet de conserver la possibilité de réaliser des travaux « de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité ».

Le projet de loi étend la procédure de réquisition de logements vacants avec attributaire à l'hébergement d'urgence, ce qui constitue à notre sens une grande avancée, alors que les besoins en la matière sont considérables en zones tendues. Le recours aux nuitées hôtelières n'est pas satisfaisant, pour les personnes hébergées comme pour les finances de l'État. La commission des affaires économiques du Sénat a réduit de deux à un an la durée de réquisition des locaux vacants à des fins d'hébergement d'urgence. Or l'atteinte au droit de propriété n'est pas disproportionnée, puisqu'il s'agit de réquisitionner des locaux appartenant à une personne morale et vacants depuis plus de douze mois, le propriétaire étant, par ailleurs, indemnisé. Dans le cadre de la mise à disposition des locaux, rien ne justifie une telle différence de régime entre les personnes sans abri et les personnes mal logées à faibles ressources, ces dernières pouvant bénéficier d'une réquisition comprise entre un an et six ans. Le présent amendement vise donc à rétablir les durées de réquisition des locaux vacants à des fins d'hébergement d'urgence telles qu'elles ont été adoptées par l'Assemblée nationale.

rédactionnelles. Sur l'amendement n° 1056 rectifié la commission a estimé que l'encadrement, dans le temps, de la réquisition, lorsqu'elle vise l'hébergement d'urgence, permet d'orienter les places de logement ainsi créées vers les populations mal logées et à faibles ressources. Cela encourage l'usage des locaux à des fins de logement, ce qui représente une solution plus durable que l'hébergement. Toutefois, il ne faut pas rallonger et renchérir les travaux par des normes superflues, sous peine de faire obstacle à la création de places d'hébergement.

en dix ans. Par cet amendement récurrent, notre groupe souhaite donner les outils pour faire de la procédure de réquisition, ouverte depuis la loi de lutte contre les exclusions de 1998, une procédure effective. Ainsi, alors qu'aujourd'hui seuls les biens de personnes morales peuvent être réquisitionnés, nous demandons d'élargir la procédure de réquisition de logements avec attributaire aux personnes physiques et aux SCI lorsque celles-ci sont détentrices d'un patrimoine immobilier de dix logements et plus. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre propriétaires à ce niveau de patrimoine. Quel est l'avis de la commission ? est l'avis de la commission ? La commission n'a pas souhaité élargir de façon démesurée le dispositif de réquisition, sous peine de remettre en cause un dispositif très stable depuis sa création en 1998, de porter une atteinte démesurée au droit de propriété et de provoquer une contraction de l'investissement locatif, et donc de l'offre de logements. L'avis est défavorable.

est d'utiliser la procédure de réquisition de locaux avec attributaire telle qu'elle existe et sans modifier les biens auxquels elle s'applique, afin de disposer effectivement d'un outil supplémentaire pour permettre l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. les locaux ciblés par la procédure seront davantage des bureaux vacants adaptés à ce type d'hébergement. Il ne me semble pas utile de procéder à une telle extension, qui pourrait

sur la recherche de solutions d'urgence se tourne vers d'autres priorités. Cette opportunité, que n'ont pas manqué de saisir les personnes morales propriétaires de biens vacants visées par cette procédure, a fait échouer toutes les tentatives de « réquisition avec attributaire depuis sa création le 31 juillet 1998. Maintenir cette disposition rendrait vaine la création de la nouvelle procédure aux fins d'hébergement d'urgence, malgré la gravité de la crise de l'hébergement et l'engagement du chef de l'État pris devant les Français le 31 décembre dernier. Cette proposition de simplification ne remet pas en cause le droit de propriété, puisque le titulaire du droit d'usage dispose de trois mois pour mettre fin à la vacance et que, dans l'hypothèse où le préfet n'a pas tenu compte de ses arguments pour abandonner la procédure, le recours judiciaire reste toujours possible. La parole

utile. Comme l'a dit mon collègue Fabien Gay, s'agissant d'une réquisition pour du logement stable, la procédure a été contournée par les personnes morales grâce à une mécanique simple : faire croire qu'elles vont faire des travaux

L'avis sera défavorable. La réquisition n'est justifiée que par la vacance prolongée des locaux, lorsque celle-ci résulte du refus du propriétaire d'y mettre fin. reviendrait, là aussi, à porter une atteinte trop importante au droit de propriété. Il est normal que le propriétaire puisse résoudre la situation soit en trouvant un usage aux locaux sous trois mois, soit en engageant les travaux nécessaires au changement d'usage. Quel est l'avis du Gouvernement émet également un avis défavorable. L'intention première de la réquisition, c'est bien le retour sur le marché locatif du logement. Aussi, il ne nous paraît pas opportun, dans l'immédiat, d'empêcher le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires à ce retour sur le marché.

le côté positif de votre démarche risque de ne pas pouvoir se mettre en oeuvre au regard de ce que je vous décris et de ce qui se produit quasi systématiquement. Les personnes morales en question connaissent parfaitement la manière de contourner les exigences qui sont celles de l'intérêt public.

Puis, dans une partie des locaux, il installe des résidents temporaires qui devront aussi s'acquitter d'une participation financière, mais également surveiller les lieux. lieux. Le résident devra respecter un règlement intérieur draconien. Par exemple, il lui est interdit de recevoir des amis, il doit laisser l'organisme inspecter son espace privé à tout moment, rentrer et quitter les lieux à une certaine heure, et ne pas s'absenter plusieurs jours sans l'autorisation de cette société

mise en place une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises de gardiennage. Il n'y a donc pas lieu de maintenir cette expérimentation à but lucratif, au bénéfice d'une société bien connue qui est aussi auteur de ce dispositif.

dans la mesure où cet amendement vise à faire évoluer le dispositif de réquisition qui est issu de l'ordonnance de 1945 en modifiant une rédaction devenue obsolète.

de manière positive ce texte en l'actualisant. Cette modification clarifie la rédaction et supprime notamment un terme devenu tout à fait obsolète et inopportun.

? L'article 12 A prévoit de prendre la date d'arrêt du projet comme date de référence pour le calcul de la consommation d'espace à dix ans. Cette date correspondant à la fin des études du diagnostic territorial, cela permettra de mieux sécuriser les procédures de SCOT. Je partage l'objectif des auteurs de l'amendement d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux procédures en cours au moment de la publication de la loi.

Cet amendement vise à offrir aux collectivités la possibilité de faire évoluer le plan local d'urbanisme une procédure de révision simplifiée lorsqu'il s'agit d'opérations de construction de logements. vigueur prévoit déjà des procédures accélérées pour faire évoluer les plans locaux d'urbanisme afin de favoriser la production de logements. La procédure intégrée pour le logement permet ainsi d'atteindre l'objectif qui est le vôtre. Elle permet de faire évoluer concomitamment

n° 145. Cet amendement vise à rétablir l'article 12 du projet de loi, qui visait explicitement la lutte contre l'étalement urbain dans les objectifs généraux du code de l'urbanisme, et qui intégrait dans les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme des actions en faveur de la densification urbaine. Alors que l'exigence de préservation de l'environnement est sans cesse réaffirmée et qu'un énième plan de sauvegarde de la biodiversité est en préparation, il semble nécessaire d'édicter des principes clairs pour guider l'action de la puissance publique.

à construire ou à rénover en milieu rural ou en bordure littorale, mais bien, dans ces zones-là comme ailleurs, de préserver le principe de continuité du bâti, et donc

partant du fait que les objectifs visés prenaient déjà largement en compte la lutte contre l'étalement urbain. Elle avait notamment cité le développement urbain maîtrisé et l'utilisation économe des espaces naturels. Par ailleurs, il ne me paraît pas utile de surcharger encore le code de l'urbanisme.

l'excellente argumentation de la sénatrice Cukierman et par les explications que vient de donner le sénateur Labbé en vue d'en revenir au texte initial. Je remercie ces deux intervenants.

explication de vote. La commission des lois a proposé à une large majorité, au travers d'un amendement, de supprimer l'article 12, et je remercie la commission des affaires économiques de nous avoir suivis, essentiellement sur l'argumentaire que vient de donner notre rapporteur Dominique Estrosi

Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait, d'un côté de l'hémicycle, ceux qui ne veulent pas consommer de terres agricoles et, de l'autre, ceux qui veulent en consommer ; ce n'est pas le sujet. Nous avons tous cet objectif de non-consommation des terres agricoles,

vote. Je veux appuyer ce qui vient d'être dit. Je suis complètement en phase avec ce qu'a dit notre collègue Joël

Cet étalement urbain conditionne aussi la crédibilité de la démarche de reconquête des zones qui sont aujourd'hui faiblement urbanisées et qui ont besoin d'être en reconversion. Le terme de densité fait peur, c'est vrai, parce que « densité » fait penser à « concentration ». Je donne souvent cet exemple, les grands ensembles créés dans les années soixante ont une densité nettement inférieure à celle de la place des Vosges à Paris.

imposent que l'on repense notre urbanisme et notre architecture. Il existe des modèles ; les Anglais ont par exemple une tendance à faire de la construction beaucoup plus dense que les Français, avec pourtant un habitat individuel très développé.

Si l'on n'agit pas sur ces questions, on aura du mal à les régler, on en restera aux bonnes intentions. Deuxième chose, il faut alléger la fiscalité sur les terres non construites-

artificialisée à 100 % est extrêmement dangereuse, car les eaux pluviales, les eaux de ruissellement, deviennent ingérables parce qu'il n'y a plus de capacité d'absorption naturelle.

pour fabriquer du carburant ou est-elle destinée à l'alimentation ? C'est une question à laquelle il faut répondre. Je ne suis pas pour que les terres agricoles fabriquent du carburant. C'est une autre approche de la société que l'on peut avoir. Je ne suivrai donc pas Joël Labbé dans son raisonnement ; je me range à l'avis de la commission.

suite à son rapport sur la fabrique de la ville. Nous avons souhaité déposer cet amendement parce que ces espaces concentrent de grandes questions d'aménagement et représentent des enjeux très importants en matière urbanistique

le plan local d'urbanisme dispose déjà des outils nécessaires pour assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. En outre, depuis le 1 janvier 2016, l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme précise très clairement que les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les principes d'aménagement des quartiers ou secteurs qui présentent des enjeux particuliers, « notamment en entrée de ville deux observations complémentaires. En premier lieu, ce plan d'aménagement spécifique aux entrées de ville constituerait un alourdissement du plan local d'urbanisme, et, eu égard à l'augmentation

l'indépendance de choix des communes et des maires, mais si, dans chaque document, on leur impose un pourcentage de telle ou telle réalisation d'équipements, je ne pense pas que cela aille dans ce sens-là.

présenter l'amendement n° 59 rectifié . Cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d'un PLU de limiter la progression des résidences secondaires. Pour favoriser la construction de logements en zone tendue, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, a supprimé les notions de coefficient d'occupation des sols et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont parfois eu pour effet de susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires. Afin d'éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées une très grande partie de l'année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures, et par un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement tend à préciser, dans le contenu du règlement du PLU, la notion de mixité sociale, en indiquant qu'en montagne elle recouvre également la question des populations saisonnières engendrées par les résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être invoquée dans le refus d'autorisation d'urbanisme lorsque le ratio des permanents par rapport aux saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable aux premiers.

Au-delà des seuls élus de la montagne, je compte sur la solidarité de tous mes collègues pour soutenir cet amendement.

J'entends bien votre préoccupation, tout à fait légitime, sur les zones à attractivité touristique forte mais saisonnière. Néanmoins, il ne paraît pas souhaitable de rattacher une telle mesure à l'objectif de mixité sociale. En outre, le critère retenu n'est pas opérationnel : l'usage d'un même bâtiment d'habitation peut changer au fil du temps et passer de résidence secondaire à résidence principale ou l'inverse. Le PLU ne peut pas figer de ratio, alors que les élus locaux n'ont pas de prise sur l'usage des bâtiments. Aussi, l'avis est défavorable.

comme résidence principale pendant une année puis comme résidence secondaire l'année suivante. En réglementer le changement d'utilisation imposerait inévitablement au propriétaire de déclarer ces changements et à la puissance publique de les contrôler.